enfin, sa responsabilité

Joël Guerriau d'avoir cosigné cet amendement. Celui-ci est gouverné par un seul objectif : garantir l'indépendance d'une commission d'évaluation pleinement opérationnelle. C'est pourquoi nous proposons des garde-fous dans les modalités de désignation et la composition de ses membres.

Comme beaucoup l'ont souligné depuis le début de l'examen de ce texte, notre APD souffre d'un grave manque de cohérence : nous soutenons des projets venant en aide aux populations, mais nous soutenons également des entreprises engagées dans des projets qui détruisent l'environnement de ces populations. Nous nous engageons à développer les économies des pays bénéficiaires de l'APD, mais nous accordons des privilèges aux entreprises françaises, pour certains projets, aux dépens des entreprises locales

afin notamment de prendre en considération les efforts déployés par les pays partenaires en vue de lutter contre la corruption et le détournement de fonds. En effet, ces efforts contribuent à prévenir toute déperdition de l'APD et méritent d'être connus,

l'évaluation stratégique de programmes et de pays- il s'agit de l'évaluation d'un ensemble d'actions, structurées pour atteindre des objectifs de développement spécifiques à l'échelle d'un secteur, d'un pays ou d'une région. Sans cet élargissement de son champ d'évaluation, la commission indépendante ne pourrait

En l'état, le texte ne spécifie pas suffisamment son mandat, alors même qu'il constitue la clé de voûte des nouveaux mécanismes d'évaluation et de redevabilité, lesquels garantissent l'efficacité et la viabilité de notre politique de développement solidaire. L'évaluation de l'efficacité de l'impact de l'aide doit, selon nous, nécessairement passer par l'évaluation du respect de la primauté des droits de l'homme, ainsi que de la cohérence des politiques publiques et de la politique de développement solidaire avec les ODD. Mes chers collègues, j'ai

cohérence. Dans le domaine agricole, nous finançons plus de projets d'agro-industrie néfastes pour l'environnement que de projets respectant nos engagements internationaux, alors que nous nous positionnons en première ligne de la lutte pour la sauvegarde de nos biens communs.

été avancé que nous n'avions pas précisé davantage les droits spécifiques reconnus à certaines populations vulnérables, quand elles seraient déjà protégées par l'inscription des droits fondamentaux. Dans les deux cas, l'exposé de nos pratiques en matière d'action extérieure démontre l'inverse. Cette commission est indispensable. Elle doit constituer un véritable outil de redevabilité et de transparence de l'APD. Pour ce faire, nous devons la doter d'un mandat clair et exigeant. Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous voterez en faveur de

qui vise à étendre le champ de l'évaluation de la commission indépendante à l'efficience des projets et programmes d'APD, afin notamment de prendre en considération les efforts déployés par les pays partenaires en vue de lutter contre la corruption et le détournement de fonds.

de prendre en considération les efforts déployés par les pays partenaires en vue de lutter contre la corruption et le détournement de fonds. Ces efforts contribuent à prévenir toute déperdition de l'APD et méritent d'être connus, pour une évaluation sans angle mort.

Enfin, nous proposons de laisser au Premier président de la Cour des comptes la charge de nommer un représentant des pays partenaires de la politique de développement solidaire.

pour objet de tirer les conséquences de l'adoption par la commission des affaires étrangères d'un amendement visant à recentrer les missions de la commission d'évaluation, créée à l'article 9. En effet, l'amendement adopté tend à préciser que la commission indépendante évalue les projets et programmes d'APD et à modifier en conséquence sa dénomination.

Au sein du présent texte, nous faisons de la dimension partenariale un principe directeur de notre politique d'aide au développement. Nous avons reconnu, et je m'en réjouis, le rôle d'expertise et la plus-value des organisations de la société civile et nous avons décidé de l'augmentation des fonds qui transitent par elles. Ce sont des avancées importantes. Toutefois, si nous reconnaissons que la mise en oeuvre ou notre aide ne peut laisser de côté la société civile, je pense que nous pouvons nous accorder sur la nécessité de l'inclure aussi dans nos mécanismes d'évaluation.

l'efficacité et l'impact de l'APD si nous prenons en compte les perspectives, les expériences et l'expertise des principaux acteurs contribuant à sa mise en oeuvre : la société civile des pays partenaires en fait partie. Les deux amendements

que les financements liés aux projets sportifs soient tracés et évalués. Cela doit permettre une meilleure connaissance et prise en compte de ces projets,

contribue à la redevabilité de cette politique, à la transparence sur les résultats atteints et à l'information du public. Le Haut Conseil à l'égalité créé en 2013, a pour mission d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l'égalité.

M. André Gattolin. Cet amendement a pour objet que la composition de la commission indépendante d'évaluation garantisse une représentation équilibrée de chaque sexe, à l'instar de ce qui est prévu

pour objet de préciser que la commission d'évaluation peut également évaluer des stratégies d'aide au développement. La mention relative à l'efficience est également pertinente, dans la mesure où il s'agit d'une question très sensible dans certains pays partenaires et où la gouvernance est encore défaillante.

sur l'amendement n° 92. Parce que la composition de la commission d'évaluation inscrite dans le texte de la commission répond pleinement aux objectifs d'indépendance et d'efficacité de cette instance, la commission émet un avis défavorable

de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les

132. L'amendement n° 299 tend à ajouter aux membres de la commission d'évaluation un représentant de la société civile des pays partenaires de la politique de développement solidaire. Or le membre représentant les pays partenaires qui est prévu par la commission pourra être issu de la société civile. La commission émet donc un avis défavorable

un avis favorable. L'amendement n° 96 a pour objet de modifier la composition de la commission d'évaluation, en remplaçant les députés, les sénateurs et les personnalités qualifiées nommées par les ministres par des personnalités qualifiées nommées par les commissions

sur l'amendement n° 288, qui tend à compléter la composition de la commission d'évaluation en ajoutant un représentant du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, désigné par son président.

à préciser que l'État et les autres personnes publiques sont tenus de répondre aux demandes d'information de la commission d'évaluation dans les meilleurs délais, la commission émet un avis favorable. n° 103 tend à préciser que la commission d'évaluation présente son rapport au Parlement, selon des modalités qui seront fixées par les deux assemblées.

exploitable et lisible par l'ensemble des acteurs des politiques de développement et qu'il soit également facilement accessible

De manière à bien appréhender cette politique, qui est extrêmement diverse, avec des champs d'application dans différentes politiques publiques,

Todeschini, sur l'article. Avec ce projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, la France a une occasion sérieuse de définir les nouveaux contours de sa politique d'aide au développement.

il s'agit tout simplement de faire du Président de la République, déjà maître des horloges, le pilote unique de l'aide publique au développement. Tous les autres acteurs sont relégués, au mieux, au rang de personnels navigants Alors que toutes nos sociétés sont traversées par de nouvelles formes de management, plus horizontales, plus transparentes, plus adaptables et plus agiles, le projet de loi prévoit la mise en place d'un conseil de développement sous l'autorité directe du Président de la République.

Ce ministre serait le responsable devant le Parlement et l'interlocuteur privilégié de tous les acteurs du développement. Plus lisible et plus démocratique, une telle méthode permettrait, par exemple, de ne plus placer les politiques de lutte contre la misère mondiale ou l'illettrisme au dernier rang des préoccupations du ministre des affaires étrangères ou dans le paragraphe perdu de quelques discours. L'aide publique au développement ne peut pas être seulement un vernis culturel pour la patrie des Lumières et des droits de l'homme. Je suis saisie

Alors que les fractures s'accroissent entre nos concitoyens et l'action politique, que la défiance entre les institutions se fait chaque jour un peu plus grande, que le contexte global est à la désinformation permanente sur fond de complotisme

illusoire : il donne à l'exécutif le sentiment de pouvoir agir rapidement, mais la précipitation n'est jamais la meilleure approche pour renforcer la démocratie. Sur l'aide publique au développement, la France a trop souvent regardé le temps court. L'heure est venue pour elle de voir plus loin, en fixant une stratégie sur le temps long. C'est d'ailleurs comme cela que cette loi a été vendue dans les médias, avant d'arriver, très tardivement, ici. Nous souhaitons donner au Gouvernement les moyens de maintenir le cap. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous opposer à la pratique du gouvernement

C'est particulièrement important au regard de l'ordonnance du 4 novembre 2020, dont nous avons longuement discuté grâce à un amendement de Mme Carlotti. Le dispositif répond à un enjeu grave, le financement du terrorisme, mais pose également de nombreux problèmes pour le secteur humanitaire. L'article 13, dans sa formulation actuelle, restreint considérablement le champ des possibles de cette évaluation, limitant l'étude d'impact à certains contextes. Cela ne permettra pas au Parlement d'envisager de manière globale l'effet de la mise en oeuvre des mesures dites « de criblage des bénéficiaires finaux tant sur l'action des organisations de solidarité internationale que sur les administrations chargées de la gestion de ces fonds. Il y a des coûts organisationnels et structurels, mais également des conséquences éthiques et de santé. Nous souhaitons donc que le rapport prenne en compte les effets des mesures de criblage sur l'action des organisations de solidarité internationale bénéficiant de financements contractuels de l'État français pour des projets de solidarité dans toute la diversité de leurs contextes d'intervention, que ce soit l'humanitaire, la stabilisation ou le développement. M. Le Drian, s'il était là, devrait tout à fait soutenir cet amendement, car il disait tout à l'heure : « La stabilisation, la zone grise, est-ce que c'est toujours de l'humanitaire ? Est-ce que c'est du développement ? On est toujours un peu hésitant. » hésitant. » Il affirmait de surcroît qu'il n'avait pas résolu ce problème de la zone grise et s'engageait à remettre un rapport sur le sujet aux commissions de nos deux assemblées. Nous souhaitons donc prévoir dans le texte que le rapport sur les mesures sur les mesures de criblage soit élargi à l'ensemble des contextes où interviennent les projets que nous finançons, afin que nous puissions juger des mesures de lutte contre le financement du terrorisme de la manière la plus informée et transparente. Quel

Sud. Je serais pour que l'on cible la politique d'aide au développement sur les 20 % de pays les plus pauvres et sur les pays à plus forte émigration vers la France ; il doit y en avoir 10 ou 15.

Ce texte, attendu depuis plusieurs années, vient concrétiser de nouvelles ambitions pour notre politique de développement solidaire, levier puissant de notre diplomatie et de notre rayonnement. Il entérine plusieurs avancées notables : une meilleure information du Parlement sur les axes de développement de ces politiques, une amélioration de la redevabilité et la création d'une commission d'évaluation des politiques de développement, même si nous regrettons que le dispositif suggéré par notre collègue Michel Canévet n'ait pas été retenu. Avec les travaux de notre commission et de notre Haute Assemblée, nous proposons un texte renforcé une meilleure hiérarchisation des priorités, avec des engagements forts, comme l'inscription de la préservation de la planète comme l'une d'entre elles, une programmation équilibrée et rallongée jusqu'en 2025, pour une meilleure crédibilité et une meilleure articulation entre les dons et les prêts de l'aide publique au développement, viennent compléter le texte. Nous nous réjouissons de l'adoption de plusieurs amendements de nos collègues membres du groupe Union Centriste tendant à favoriser l'apprentissage du français et la francophonie, outil indispensable de notre rayonnement à l'international. La reconnaissance des outre-mer comme véritable atout stratégique, le soutien à nos entrepreneurs à l'étranger et les politiques en faveur des droits des enfants nous paraissaient également indispensables, et nous nous félicitons de l'adoption de nos amendements sur ces sujets. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste

À bien des égards, le Gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique et de son ambition, pourtant annoncées dès le début du quinquennat. C'est particulièrement le cas en matière de programmation financière, puisque la trajectoire nous a été présentée tronquée et sans objectifs chiffrés. C'est grâce au Sénat que nous sommes passés du virtuel au réel, avec une proposition ambitieuse : la taxe sur les transactions financières sera désormais fléchée à hauteur de 60 %, au lieu de 30 %, pour l'APD.

Nous avons finalisé le mécanisme de restitution des biens mal acquis. Le groupe SER a proposé qu'un article soit dédié à l'obligation de vigilance ; il nous paraissait normal que nos entreprises aient un comportement éthique et que, par extension, lorsqu'elles constatent des manquements, elles soient tenues de les signaler à la justice. Vous n'en avez pas voulu complètement. C'est regrettable, d'autant qu'il s'agit d'un recul significatif par rapport à la loi de 2014. Sachez que nous resterons extrêmement vigilants sur le ciblage de l'APD en direction des 19 pays prioritaires, particulièrement ceux du G5 Sahel. C'est une nécessité absolue absolue pour venir en aide aux populations et soutenir l'action de nos troupes dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons voulu mettre l'accent sur les enjeux de santé. Nous ne sommes pas parvenus à obtenir la levée des brevets, mais nous sommes convaincus que, sous la pression de l'opinion publique mondiale, la France s'alignera sur cette position. cette position. pour la participation de la France au fonds dédié à la constitution d'états civils fiables dans les pays les plus pauvres. Nous avons obtenu la reconnaissance des populations précaires et mis l'accent sur l'extrême pauvreté. Nous aurions voulu aller plus loin sur les droits sociaux et sur les services publics de base, notamment l'éducation ; là aussi, la loi de 2014 était beaucoup plus progressiste. Mais nous avons obtenu des avancées, considérables, sur les questions de genre. Mes chers collègues, le débat fut long, respectueux et, quelquefois, assez riche.

flou : malgré notre insistance, un grand silence demeure sur la cohérence d'ensemble de nos politiques. Nous risquons donc de continuer à donner d'une main ce que nous reprenons de l'autre à travers les conventions fiscales, les politiques commerciales

Le projet de loi que nous allons voter n'est pas parfait, mais il a le mérite de poser de nouveaux éléments fondamentaux, tels que le pilotage stratégique et politique des acteurs de l'aide publique au développement. Notre

N'oublions pas que l'aide publique est un levier d'influence nécessaire à notre pays, face à l'agressivité des nouveaux pays émergents, qui font de l'aide sans nos valeurs.

les fameux 0,7 % de notre richesse nationale à l'aide publique au développement. Nous n'y sommes pas, hélas ! Toutes les propositions qui auraient permis d'améliorer, et surtout de sécuriser notre programmation ont été rejetées.

sommes déçus de constater que nous ne voulons pas renforcer le devoir de vigilance dans notre action extérieure, alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, en 2017, déjà trois de nos grandes entreprises multinationales sont devant la justice. Les acteurs publics et privés à l'étranger ont une haute responsabilité ; ils doivent impérativement changer leurs pratiques, pour ne pas miner les succès de notre aide publique au développement. À ce titre, si nous nous réjouissons des avancées que porte ce texte sur d'autres questions, nous regrettons qu'il ne prévoie pas plus de transparence et de contrôle de l'action de nos acteurs publics et privés à l'étranger et qu'il n'ait pas reconnu le besoin de rechercher activement une cohérence entre notre politique d'aide et les autres politiques ayant un impact sur les aidées. Nous conserverons donc un regard particulièrement vigilant sur notre politique d'aide au développement. Nous reconnaissons cependant, avec plaisir, les acquis de ce texte et l'apport du Sénat, notamment sur la promotion et le respect des droits humains, en particulier le droit des enfants, des femmes, des filles et des peuples autochtones, sur le renforcement relatif de nos moyens d'aide au développement, avec l'extension de la programmation, sur le principe de non-discrimination en zone de guerre, sur la reconnaissance d'un certain nombre de conventions internationales